nationale, que des arbitrages avaient été rendus et que la ministre, Mme Buzyn, avait obtenu certaines concessions de la part du Premier ministre concernant, en particulier, la reprise de la dette des hôpitaux ou l'évolution de carrière des professionnels

que notre pays décide d'assigner à notre système de santé pour les cinq années à venir et des moyens à lui affecter pour répondre à ces objectifs.

là où c'est nécessaire- on le sait, l'hôpital a perdu en vingt ans 100 000 lits -, revaloriser les salaires, rendre plus attractives toutes les professions à l'hôpital, stopper la fuite des professionnels, investir dans la psychiatrie, parent pauvre de notre système de santé, investir pour l'avenir dans l'immobilier hospitalier, les équipements et l'innovation. Quel est l'avis de

pour que les tarifs 2020 soient au minimum aussi bons, voire en amélioration par rapport à ceux qui ont été pratiqués en 2019. Vous le savez, nous travaillons à un plan global pour l'hôpital, qui vise à renforcer nos capacités d'investissement, notamment dans le quotidien

sur trois ans, des tarifs hospitaliers. Nous étudions évidemment toutes les mesures qui permettront de restaurer de la marge de manoeuvre à l'hôpital public et de rendre plus attractives les carrières, mais cela ne nécessite pas une loi d'orientation particulière.

ne serait-ce que parce qu'il faut que nous sachions exactement où nous allons par rapport aux hôpitaux. Si, dans le cadre de la nouvelle lecture, les propositions faites par la ministre sont satisfaisantes, le rapport n'aura plus lieu d'être. En attendant, nous souhaitons mettre un peu la pression sur le Gouvernement pour l'inciter à nous présenter un rapport acceptable.

ministre, les mesures que vous avez dégagées jusqu'à présent sont loin d'être suffisantes compte tenu de la situation réelle de l'hôpital. La preuve en est : les services d'urgences et, au-delà, l'ensemble des hôpitaux sont en lutte, toutes professions confondues, depuis huit mois. Les manifestations qui vont avoir lieu dans quelques jours prouvent la colère et l'amertume des professionnels de santé.

inconvénient. Du point de vue de la justice sociale et de la solidarité, il en va tout autrement. Je dois rappeler ici que le budget de l'État est financé en grande partie par l'impôt sur le revenu, alors que le budget de la sécurité sociale est financé par les cotisations sur le travail.

Pour 2020, le déficit prévisionnel est à peine réduit à 5,1 milliards d'euros. Certes, la masse salariale est moins favorable que prévue, certes les dépenses des branches maladie et vieillesse sont plus élevées qu'attendues, mais, surtout, les mesures adoptées dans le cadre de la loi Mesures d'urgence, en décembre dernier, pèsent pour près de 2,7 milliards d'euros et ne sont pas compensées par le budget de l'État. En refusant de compenser par les crédits du budget de l'État les conséquences de ses propres choix fiscaux, le Gouvernement déroge à la loi Veil de 1994, qui avait instauré une sorte de règle d'or- le président

intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État ». Vous organisez- le terme a déjà été utilisé -une sorte de pillage de l'édifice social issu des ordonnances de de 1945, qui est non pas le produit d'un monde ancien, mais un édifice de valeurs : la solidarité, la justice, dont découle l'autonomie de la sécurité sociale. À l'aube du retour à l'équilibre de la sécurité sociale, Bercy- c'est ainsi que l'on s'exprime -fait peu de cas de son autonomie, accroît son emprise et prépare la captation des excédents potentiels des années suivantes. Comment ne pas percevoir l'orchestration politique de ce déficit, pour le déplorer et pouvoir poursuivre une politique d'austérité ? Quelle sera la prochaine étape ? La fongibilité totale du budget de l'assurance maladie dans celui de l'État ? Hier, il nous a été indiqué que cette perspective n'était pas réelle ; nous osons l'espérer ... La parole

le problème des hôpitaux ; c'est en tout cas ce que vous venez de nous dire. Nous pensions que les décisions étaient déjà prises, qu'il y aurait une réponse construite aux difficultés des hôpitaux,

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. » L'article 3 du PLFSS pour 2020 propose, quant à lui, que ce crédit d'impôt ne fasse pas l'objet d'une compensation à la sécurité sociale. Or les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l'État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale », défini à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. De plus, cette politique d'exonération de cotisations sociales a des conséquences directes sur le financement de notre système de protection sociale, fondé sur la solidarité et la collectivité. Par ailleurs, la Cour des comptes relève, dans son dernier rapport, un déséquilibre des comptes de la sécurité sociale, qui s'explique, avant tout, par la politique d'exonération de cotisations sociales. C'est la raison pour laquelle il est proposé, au travers de cet

de celui-ci, vous vous apprêtez à prendre une décision grave pour notre système de sécurité sociale : vous amputez son budget de plus de 3 milliards d'euros alors que vous ne cessez de mettre en avant un déficit de 5 milliards

l'exception au principe, c'est ce que vous êtes en train d'acter, en prévoyant la non-compensation, par l'État, des mesures dites « gilets jaunes », qui coûtent plus de 3 milliards d'euros à la sécurité sociale.

Quelles en seront les conséquences pour nos concitoyens ? Des coupes budgétaires sur les hôpitaux, avec fermetures d'établissements publics, de services, de lits, et des Ehpad sinistrés ! Quel signal envoyez-vous à l'ensemble de la population ? Les faibles primes accordées à quelques-uns ne suffiront pas à compenser la facture de la casse du service public de la santé. Quel

par le principe de « compensation intégrale », défini à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Ce principe a été respecté pendant le précédent quinquennat, mais, depuis 2017, des entorses à cette règle ont été observées, comme le crédit d'impôt de taxe sur les salaires, qui n'a pas fait pas l'objet d'une compensation à la sécurité sociale en 2018. Pour 2020, ces non-compensations à la sécurité sociale s'élèveraient à un montant estimé à 3,5 milliards euros : 1,2 milliard d'euros d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 1,5 milliard d'euros de baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 euros par mois et une diminution de 800 millions d'euros sur le forfait social. Par conséquent, l'article 3 prive la sécurité sociale de 3,5 milliards d'euros de ressources qui devaient lui revenir. Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas de l'article relatifs à cette non-compensation.

Le Gouvernement doit entendre que la compensation, par l'État, de mesures d'exonérations sociales est bien le principe et non l'exception. Il n'a pas à financer les choix politiques de l'État par l'argent des assurés sociaux. Il est de la responsabilité de l'État de financer ses propres politiques. Par ailleurs, c'est un non-sens absolu que de demander aux assurés sociaux de financer eux-mêmes l'augmentation de leur pouvoir d'achat, sans parler des travailleurs et travailleuses qui n'ont pas bénéficié des mesures d'urgence économiques et sociales ; ceux-ci paient les frais d'une mesure qui ne les concerne pas ! En effet, la prime est facultative ; la loi n'oblige pas les entreprises à verser cette prime à leurs salariés, il s'agit seulement d'une incitation. L'objet de cet amendement est de revenir non sur la nature des mesures prises, mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.

versant de l'intéressement ou de la participation, mesure décidée dans le cadre de la loi Pacte, et qui engendre une perte de recettes de 500 millions d'euros. Monsieur le secrétaire d'État, même si, depuis le vote de la loi Veil, il y a eu d'autres exemples

Elle s'oppose au principe, posé par la loi Veil en 1994, selon lequel « toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État. » des interrogations sur les marges de manoeuvre réelles dont nous disposons, alors que deux échéances cruciales sont encore devant nous. D'une part, le grand chantier de la dépendance nécessitera un besoin de financement public supplémentaire de l'ordre de 6,2 milliards d'euros à 2024 et de 9,2 milliards d'euros d'ici à 2030. C'était tout l'objet des propositions du rapport, de Dominique Libault, ancien directeur de la sécurité sociale et actuel président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Face au défi majeur du vieillissement de la population, ce rapport apportait des réponses claires et ambitieuses aux inquiétudes des Français sur l'accompagnement de leurs vieux jours.

système de retraite. On craint, en particulier, que la rupture avec le principe de non-compensation ne conduise le Gouvernement à faire supporter par la sécurité sociale le financement des régimes de retraite de la fonction publique, qui sont aujourd'hui du ressort de l'État. Cet amendement vise donc à revenir sur la non-compensation des mesures décidées au travers de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales : la baisse de la CSG pour les retraités, avec la création d'un taux intermédiaire, et l'avancement de l'exonération sur les heures supplémentaires.

l'État compense très largement les exonérations que supporte la sécurité sociale ; je pense aux allégements généraux financés par l'affectation d'une fraction de TVA, à hauteur de plus de 51 milliards d'euros. En outre, nous assumons bien évidemment le fait de demander à la sécurité sociale de financer

1 milliard d'euros non compensés par l'État à la sécurité sociale- c'était donc déjà une somme importante. Tout cela pour rappeler aux uns aux autres que ce principe n'a pas toujours été respecté. Nous avons la conviction que

notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales, qui met en péril notre système collectif de protection sociale. Les magistrats de la Cour, que l'on ne peut pas qualifier de « révolutionnaires », vous en conviendrez, mes chers collègues, indiquent indiquent que « la place aujourd'hui acquise par les allégements généraux de cotisations qui bénéficient à l'ensemble des employeurs de salariés interroge la définition même de la norme de référence en fonction de laquelle des règles particulières sont qualifiées de dérogatoires ». écologiste, la priorité pour financer la sécurité sociale doit être de supprimer les exonérations de cotisations, de rétablir les cotisations à l'ensemble des branches de la sécurité sociale, de lutter contre la fraude patronale et de mettre à contribution les revenus financiers et les industriels pharmaceutiques, qui profitent très largement de notre système de protection sociale. Une fois ces mesures adoptées, nous pourrons moderniser le principe fondamental selon lequel chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins.

D'après l'Observatoire des inégalités, en 2016, les 10 % des salariés les moins bien rémunérés touchent au mieux 1 200 euros par mois, quand le club du 1 % des salaires les plus élevés gagne plus de 8 600 euros Pour ces raisons, nous proposons, au travers de cet amendement, de relever les cotisations sociales sur les plus hauts salaires. En effet, aujourd'hui, les hauts salaires cotisent au même niveau que les salaires les plus bas. La solidarité nationale est la base de notre contrat social, elle doit être rétablie. Les personnes aux revenus les plus élevés doivent y contribuer ; c'est une question de justice sociale.

contrevient au principe d'égalité devant l'impôt, dans la mesure où il vise à déterminer un taux de cotisation en fonction de la nature d'un revenu et non de la capacité contributive du foyer fiscal.

la multiplication des exonérations de cotisations sociales met en péril notre système de protection solidaire. Alors que le niveau des exonérations et allégements de cotisations a dépassé les recettes de la branche famille, famille, nous proposons, au travers de cet amendement, de redéfinir les relations entre l'État et la sécurité sociale. Selon nous, la seule doctrine qui vaille, c'est de dire « stop

pourquoi nous proposons un mécanisme démocratique visant à verrouiller la prolifération des exonérations de cotisations sociales. En effet, la sécurité sociale appartient aux assurés sociaux et à leurs représentants, et à leurs représentants, au travers de la gestion paritaire par les syndicats et le patronat. Il est inadmissible que les décisions qui ont des conséquences aussi graves que la non-compensation des exonérations par l'État entraînent un déficit et donc réduisent les prestations des assurés sociaux. Pour toutes ces raisons, nous proposons que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fasse l'objet d'un vote de la part des caisses de sécurité sociale. Quel

pour dire que la création d'un pôle public du médicament serait à même de mettre un terme aux ruptures de stock organisées par les industriels. Tant que notre pays ne retrouvera pas la capacité publique de produire et de distribuer des médicaments, les industriels resteront libres de stopper la production des médicaments dont le taux de rentabilité est décroissant.

pour financer un véritable pôle public du médicament qui permettrait au Gouvernement de reprendre la main. Aujourd'hui, le Gouvernement n'a pas la possibilité d'imposer à tel ou tel grand laboratoire la production

Au prétexte que le chiffre d'affaires de la filière industrielle aurait diminué en 2018, vous décidez, madame la ministre, de relever le taux à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche de 0,5 % à 1 %. Mais vous oubliez de rappeler que, en 2017, le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en France avait augmenté de 14 %, passant à 43 millions d'euros, après dix ans de résultats stables. Dès lors, l'année 2018 a marqué non pas une baisse, mais un retour à la normale après une année exceptionnelle en matière de résultats. Surtout, en relevant le taux à partir duquel l'industrie contribue à la sécurité sociale, vous privez une nouvelle fois de recettes supplémentaires notre système solidaire cette baisse de 60 millions d'euros pour la sécurité sociale en 2019 aurait pu utilement servir au financement du service public hospitalier. En outre, ce cadeau paraît injustifié au moment où certaines entreprises du médicament, bien portantes financièrement, licencient massivement dans notre pays. Je pense notamment au groupe Sanofi, qui prévoit actuellement un plan social de 300 personnes, malgré un bénéfice net de 6 milliards d'euros en 2018 et après avoir touché 300 millions d'euros de crédit d'impôt. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 4.

Apourceau-Poly, sur l'article. Pour l'année 2019, l'objectif d'amortissement de la Cades était fixé à 16 milliards d'euros. Ce sont donc 16 milliards d'euros qui sont allés au remboursement de la dette plutôt qu'au financement de prestations, notamment dans les hôpitaux publics. Je rappelle que la dette de la sécurité sociale, remboursée à marche forcée, provient du transfert, dans les années 1980, des bons du Trésor vers les marchés financiers, qui ont demandé un taux de rendement extrêmement élevé. Nous contestons l'objectif

Alors que le Gouvernement songe à reprendre 30 milliards d'euros de la dette des hôpitaux, nous devons poser la question de la légitimité de la dette, issue de créances d'établissements privés à taux variables ou extrêmement défavorables

rendant les conditions de travail extrêmement difficiles. Même la meilleure organisation des services qui soit ne peut fonctionner infiniment sans atteindre ses limites, à partir du moment où ses problèmes ne sont pas réglés et où des moyens supplémentaires ne lui sont pas accordés.

Comme l'intersyndicale et le collectif Inter-Urgences, nous demandons 10 milliards d'euros supplémentaires en 2020, ce qui correspond à l'évolution naturelle des dépenses, avec un Ondam à 4,5 %.

Cette situation de tension, que l'on retrouve dans les Ehpad, mais aussi dans les services accueillant des personnes en situation de handicap, est le fruit d'une politique austéritaire ainsi que d'une pression mise sur les finances de la sécurité sociale. Les propositions faites au travers du présent PLFSS ne sont pas à la mesure des enjeux. Les dépenses relatives aux établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes à l'heure où l'hôpital public est en très grande difficulté.

habitude. Les Français savent pertinemment que notre hôpital est en train de mourir de cette rigueur budgétaire aveugle qui s'est renforcée au cours du temps.

et la pénurie de l'hôpital public

officiellement devant vous. L'affaire est donc réglée. Il est hors de question aujourd'hui de proposer à la vente des hôpitaux publics : les hôpitaux publics resteront dans le giron du secteur public hospitalier.

En reconduisant le dispositif de la prime exceptionnelle, avec exonération de cotisations sociales, le Gouvernement, soutenu par le patronat, souhaite tout simplement éviter la généralisation et l'amplification du conflit social dont les « gilets jaunes » ont été le moteur voilà un an, tout en préservant les intérêts capitalistes. En effet, cette mesure faussement en faveur du pouvoir d'achat contourne la revendication juste et légitime des travailleurs et travailleuses de ce pays d'une augmentation générale des salaires et des pensions. Le patronat des grandes entreprises, puisque ce sont elles qui ont majoritairement mis en place ce dispositif, préfère bien évidemment verser quelques miettes plutôt que de subir un mouvement social d'une ampleur inédite risquant de remettre en cause ses intérêts financiers. Et comme si le mépris du Gouvernement à l'égard des revendications des travailleurs n'était pas déjà insupportable, ce dernier en rajoute une couche en privant la sécurité sociale des cotisations patronales, ce qui creuse encore son déficit. Encore une fois, ce dispositif est la preuve éclatante de l'organisation du déficit de la sécurité sociale par le Gouvernement.

1 000 euros. Cette mesure a rencontré un franc succès, comme le prouvent les chiffres enregistrés : 5 millions de salariés en auraient bénéficié entre fin 2018 et début 2019 pour un gain moyen de 400 euros. C'est donc naturellement que ce projet de loi reconduit cette mesure pour

de nombreuses entreprises n'ayant pas la capacité financière d'associer leurs salariés aux résultats ou aux performances. Nombre de salariés pourraient s'en trouver

408 000 d'entre elles auraient versé cette prime à près de 5,5 millions de salariés, pour un montant moyen de 400 euros. Subordonner son versement à l'existence d'un accord d'intéressement risque,, d'exclure du dispositif

cotisations sociales. Accorder cette prime aux grandes entreprises apparaît injuste, car elles ont la capacité d'augmenter les salaires sans passer par des dispositifs dérogatoires exonérés de cotisations sociales. En outre, ces grandes entreprises sont aujourd'hui les principales utilisatrices des dispositifs d'intéressement, qui leur permettent de verser des primes à leurs salariés sans régler les cotisations sociales obligatoires. Ainsi, l'intéressement bénéficie à hauteur de 75 % aux employés des entreprises de plus de 1 000 salariés. À l'inverse, la prime peut se justifier pour les plus petites entreprises, qui utilisent encore peu l'intéressement, malgré l'exonération de forfait social décidée dans le cadre de la loi Pacte. Cet amendement de repli

et 576. Toutefois, plus la prime exceptionnelle sera dérogatoire et inconditionnelle, plus grand sera le risque de la pérenniser, au détriment des finances de la sécurité sociale. la sécurité sociale. Dans l'intérêt même des salariés et de leur pouvoir d'achat, il serait utile de profiter de cette prime pour promouvoir l'intéressement dans le plus grand nombre d'entreprises.

pour un montant moyen de 1 700 euros par an, ce qui est loin d'être négligeable. C'est la raison pour laquelle nous proposons que le bénéfice de la nouvelle prime, intégralement défiscalisée et reconduite en 2020, soit subordonné à la mise en place d'un accord d'intéressement, avant le 30 juin 2020, pour toutes les entreprises. Par rapport à la prime exceptionnelle, l'accord d'intéressement et de participation est plus avantageux : aucune taxe pour les entreprises de moins de 250 salariés, puisque nous avons supprimé le forfait social depuis le 1 janvier 2019 2019 ; aucune taxe pour les salariés non plus, puisque les sommes sont épargnées- mais rien n'empêche le salarié de bénéficier immédiatement des sommes versées, alors fiscalisées ; contrairement à la prime, l'accord apporte une visibilité sur plusieurs années- jusqu'à trois ans -, même s'il sera exceptionnellement possible de le conclure pour un an seulement, en 2020 ; enfin, et nous rejoignons là une des préoccupations de M. le rapporteur général, l'accord permet d'éviter les effets d'aubaine et constitue une garantie contre la substitution de la prime au salaire.

suffise à la mise en oeuvre de ces accords. Nous sommes convaincus que l'accord d'intéressement apporte de la stabilité et qu'il permet de mettre en place des dispositifs de partage de la valeur créée dans les entreprises de manière plus pérenne que la seule prime exceptionnelle. Pour ces raisons, le

mais un outil de captation du salaire socialisé, qui peut engendrer une diminution de la masse salariale, donc des perceptions de cotisations sociales pour la sécurité sociale. Son octroi diminue les droits à la retraite des salariés et le droit au chômage et ne contribue pas au financement du système de santé, à l'assurance maladie, aux retraites et aux hôpitaux, à un moment où ils en ont éminemment besoin. Facultative pour les entreprises, cette prime masque d'autres enjeux plus importants, comme l'augmentation du SMIC, des minima sociaux ou encore du point d'indice de la fonction publique. Je veux le souligner, l'Acoss a relevé un repli de la masse salariale de 0,3 % pour le premier trimestre de 2019, après une augmentation de 0,8 % au cours du dernier trimestre de 2018. Sans doute parce que les entreprises ont versé une prime en 2018 et procédé ensuite à une compression salariale pour amortir leurs dépenses. L'Insee conforte d'ailleurs cette analyse dans une note de conjoncture publiée au mois de mars. La parole

l'attitude des salariés qui en ont bénéficié. J'ai utilisé ces termes en écho à un point de convergence que nous avons avec M. le rapporteur général sur le fait que cette prime exceptionnelle ne doit pas avoir comme conséquence de se substituer aux salaires, pour les raisons qui ont été évoquées. Une partie d'entre elles ont été rappelées par M. Daudigny à l'instant, d'autres ont été rappelées par M. le rapporteur général. Cette prime est un succès. Nous souhaitons la reconduire, en lui donnant une forme de pérennité et de stabilité,

le côté pratique de ces outils, mais je puis vous assurer que nous avons veillé à ce qu'ils soient aussi pratiques et maniables que possible. Les accords types permettent véritablement à toutes petites entreprises

à l'occasion de l'examen de la loi Pacte. Il s'agissait de fixer des objectifs en matière de développement et de progression du nombre d'accords d'intéressement et d'accords de participation.

et la loi de finances rectificative que vous aurez bientôt à examiner tend à ajouter 800 millions d'euros supplémentaires pour financer l'augmentation des dépenses en matière de prime d'activité. L'Insee l'a souligné, 2019 restera comme une année de progression majeure du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français, avec des taux de progression qui n'avaient pas été atteints depuis plus de dix ans. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.

il s'agit d'exclure la condition de mise en oeuvre d'un accord d'intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les établissements privés à but non lucratif du champ sanitaire, social et médico-social. Dans les faits une très faible part de ces établissements l'a mise en place. Or, compte tenu des revenus, souvent faibles, dans ces établissements et des difficultés rencontrées au cours rencontrées au cours des dernières années et plus particulièrement en ce moment, ainsi que des efforts importants consentis par les salariés, permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette prime exceptionnelle apparaîtrait comme un geste notable en faveur du pouvoir d'achat

de la commission ? Cet amendement est intéressant, mais il n'est pas rédigé conformément à son objet. En cas d'adoption, les établissements visés ne pourront tout simplement pas verser la prime exceptionnelle, qu'ils aient ou non conclu un accord d'intéressement.

Mais vous passez sous silence un élément important : vous supprimez la partie socialisée du salaire, celle qui permet une sécurité face à la maladie, un soutien matériel et financier pour la famille, une garantie d'avoir une retraite digne de ce nom. C'est très pernicieux. Prenons un autre exemple, celui de votre mesure visant à supprimer les cotisations des salariés pour l'assurance chômage. Certes, le résultat immédiat est un gain du pouvoir d'achat, avec un salaire net légèrement supérieur. Mais quelle est la conséquence de la suppression des cotisations d'assurance chômage ? Une baisse des indemnités chômage pour des centaines de milliers de chômeuses et chômeurs et un durcissement des règles d'ouverture de leurs droits. Et la situation va s'aggraver, puisque vous allégez également les cotisations patronales pour l'assurance chômage ! C'est en quelque sorte un miroir aux alouettes : il ne faut pas regarder

bien accueillie par les salariés, même si elle ne bénéficie pas à tous, comme cela a déjà été indiqué. Nous l'avions d'ailleurs voté l'an passé, dans des conditions elles-mêmes exceptionnelles. Il convient, Il convient, nous le pensons, de rétablir les cotisations et contributions sociales, afin de ne pas amputer le budget de la sécurité sociale d'une partie de ses recettes. Il faut le souligner, ces cotisations et contributions permettent également d'augmenter les droits des salariés. La prime exceptionnelle ne doit pas devenir la règle, au détriment des mesures de salaire. L'amendement vise à contribuer à prévenir ce comportement, par la mise en oeuvre d'une solution équilibrée consistant à défiscaliser mais à ne plus désocialiser la prime. Quel soumise à l'ensemble des cotisations et contributions sociales. Ils ont le mérite de souligner qu'il ne serait guère supportable, c'est ce que vient de dire Yves Daudigny, pour les finances sociales, de pérenniser ce dispositif, année après année.

le fonctionnement de notre service public de santé ... La réalité, c'est que nous ne nous donnons pas les moyens d'avoir une protection sociale à la hauteur des besoins et des attentes de nos concitoyens.

une cotisation comparable à la CSG, c'est-à-dire une contribution additionnelle. Ce serait bien plus juste que l'augmentation de la CSG pour les retraités, en particulier les retraités modestes

le Sénat avait obtenu, en commission mixte paritaire, la mise en place d'un stage obligatoire en autonomie d'au moins six mois pour les étudiants en médecine de troisième année de troisième cycle.

Bien que nous soyons opposés à la politique d'exonérations sociales, nous pensons que celle-ci peut être utile pour la collectivité lorsqu'elle permet une réelle avancée en matière de conditions de travail L'objectif du dispositif que nous défendons est de montrer que les salariés travaillent mieux et sont en meilleure santé lorsqu'ils travaillent moins. Cela a nécessairement un impact positif sur l'entreprise comme sur les caisses de la sécurité sociale. Par ailleurs, la réduction du temps de travail à 32 heures permettrait de réduire très rapidement le chômage par la création de millions d'emplois, en plus de redistribuer les richesses de manière plus équitable. Aussi, les employeurs jouant le jeu seraient récompensés en étant exonérés de cotisations patronales sur les contrats à durée déterminée conclus dans ce cadre. En adoptant notre amendement, mes chers collègues, nous montrerions qu'il est possible d'opter pour une autre philosophie en matière d'exonérations sociales, en subordonnant celles-ci à des comportements vertueux. Quel